La séance est ouverte,

qui j'aurai la parole dans quelques instants, s'il y a pas d'autres observations le procès verbal est adopté sous les réserves d'usage. Mise au point, je le président Claude Malhuret, président du groupe, les indépendants, République et Territoires souhaité faire une mise au point sur un vote.

Acte de cette demande Madame Nicole Duranton. Merci Monsieur le Président, rectification de vote également sur le scrutin, numéro 120 sur l'article 2 du projet de loi maintenant provisoirement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre la Covid 19 Marie-Laure Phinera Horth souhaitent s'abstenir. Nous donnons acte cette mise au point ces de mise au point, seront publiés au Journal officiel et figureront dans l'analyse politique du scrutin. L'ordre du jour, mes chers collègues, appelle la discussion du projet de loi autorisant la ratification du protocole au traité de l'Atlantique nord sur l'accession de la République de Finlande et la ratification du protocole ou même traité sur l'accession dure une royaume de Suède la procédure accélérée a été engagée sur ce texte dans la discussion générale, je vais donner la parole à Madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe. Et des Affaires étrangères, madame la ministre.

Merci monsieur le président, monsieur le président, monsieur le rapporteur, c'est le président Combo mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs, je suis honoré de présenter aujourd'hui au Sénat, le projet de loi visant à autoriser la ratification des 2 protocole au traité de l'Atlantique nord sur l'accession de la République de Finlande et du royaume de Suède. Vous mesurez comme moi je le sais, l'importance de ces deux textes et je tiens à vous remercier d'avoir permis leur examen rapide malgré l'agenda particulièrement lourd, qui est le vôtre, les demandes d'adhésion formulée par Stockholm et par Helsinki constituent une évolution historique pour ces 2 pays attachés traditionnellement à des politiques de non participation à des alliances militaires pour la Suède, il s'agit d'une rupture avec près de 2 siècles d'une neutralité décidé suite au conflit qui avait opposé la Suède et la Norvège en 1814 pour la Finlande cette décision tourne la page des premières heures de la guerre froide et de la neutralité forcée imposée par l'Union soviétique en 1948. Difficile à envisager, il y a encore 6 mois, ces demandes sur la conséquence directe de l'évolution de notre environnement de sécurité provoquée par l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine depuis le 24 février. Ces demandes sont le fruit de décisions souveraines prise à l'issue d'importants travaux de consultation nationale et internationale, reflétant des évolutions majeures de l'opinion publique dans chacun de ces 2 pays, je signale au demeurant que la Finlande et la Suède avait déjà adapté leur politique de défense, à la suite de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation du Donbass en 2014 et plus généralement dans le contexte marqué par une posture russe, de plus en plus menaçante et de plus en plus agressive, c'est demanderai un besoin de sécurité accrue de la Suède et de la Finlande en devenant les 31ème et 32ème Membre de l'Alliance Atlantique, ces 2 alliés pourront bénéficier du principe fondateur de l'Alliance, qui est l'obligation d'assistance en cas d'attaque armée contre l'un de ses membres. Obligation inscrite à l'article 5 du traité de l'Atlantique nord, ces adhésions constitueront également un gain pour la sécurité de l'espace Baltique et pour la sécurité collective des Européens, en effet, la Suède comme la Finlande dispose de capacités militaires robuste qui contribueront significativement à la sécurité de l'ensemble des alliés. L'armée finlandaise compte parmi les plus fournies d'Europe en matière d'effectifs et d'artillerie, la Suède, qui entretient une industrie de défense compétitive ah non, a annoncé de son côté une importante revalorisation de son budget de défense pour atteindre bientôt les 2 % du Toutes 2 sont dotées de capacités et d'équipements qui sont déjà communs de nombreux alliés permettant ainsi une parfaite interopérabilité au sein de l'OTAN, je suis navré en doute que la France a pu voir à l'oeuvre et apprécié des capacités suédoise et finlandaise dans le cadre de la participation active d'Helsinki et de Stockholm à la politique de sécurité et de défense commune de l'Union Européenne dans des zones prioritaires pour nos intérêts la Suède notamment activement construit buée à la Task Force Takuba de 2020 cette année au Sahel et depuis 2013 à la Mission intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali, la Minusma. De son côté, la Finlande, participe à la mission de formation de l'Union européenne au Mali EUTM Mali et à la Minusma. Par ailleurs, l'engagement, ces 2 pays pour la défense européenne ne fait aucun doute, en témoigne leur participation à l'initiative européenne d'intervention dite une une dont la principale vocation est de faire émerger une culture stratégique et opérationnelle communes aux Européens. Enfin, et c'est un point fondamental : l'adhésion de la Suède, la Finlande, renforcera la place des Européens dans l'Alliance Atlantique en portant à 23 le nombre d'États de l'Union européenne au sein de l'Alliance ces adhésions consoliderons l'OTAN elles-mêmes mais aussi son pilier européen. Cela aura également un effet bénéfique pour l'autonomie stratégique de l'Union Européenne, c'est-à-dire sa capacité à assurer elles-mêmes la défense de ses propres intérêts de sécurité, c'est d'ailleurs une ambition de plus en plus assumé par ses États comme le montre la décision récente du Danemark, soutenu par voie de référendum par plus de 66 % de sa population, de s'intégrer désormais pleinement à la politique européenne de sécurité et de défense commune. L'adhésion de la Suède et de la Finlande confortera en outre les choix stratégiques faits par de nombreux États membres qui, à la suite notamment du sommet de Versailles en mars dernier, ont décidé de réinvestir dans leur défense et je précise qu'il ne s'agit pas de compétition entre organisations mais bien d'un vaste mouvement de réveil stratégique de la part de nos partenaires, mouvement qui bénéficiera total, autant que l'Union européenne à notre sécurité collective européenne et transatlantique et donc à la sécurité de la France et des Français. Pour l'ensemble de ces raisons, monsieur le rapporteur, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, il est fondamental que nous soyons au rendez-vous de ce mouvement de ce moment historique pour la sécurité européenne. C'est notre responsabilité et c'est notre responsabilité, à plusieurs égards. Tout d'abord vis-à-vis de l'ensemble de nos alliés, dont les chefs d'État ou de gouvernement ont soutenu à l'unanimité, les candidatures de Stockholm et d'Helsinki lors du sommet de l'OTAN à Madrid le 29 juin dernier. Comme vous vous en souvenez, cette unanimité a été difficile à obtenir en raison des réserves d'un allié de la Turquie au motif affiché de différends bilatéraux, en particulier avec la Suède, concernant la lutte contre le PKK. Ces réserves ont été levées, à la faveur d'un mémorandum d'entente avec la Finlande et la Suède, conclu par la Turquie, avec ces 2 pays en marge du sommet, je précise cependant que si ce mémorandum a eu le mérite de lever les réserves turc, il ne constitue en rien un engagement de nature alliés de l'OTAN, ni l'ensemble de ses membres. Cet accord a ouvert la voie le 5 juillet à Bruxelles à la signature des protocoles d'adhésion par la Suède, la Finlande, ainsi que les représentants permanents des 30 alliés auprès de l'OTAN, la phase de ratification par les 30 alliés selon le droit interne de chacun est ouverte depuis lors, plusieurs d'entre eux ayant eu recours à des procédures accélérées ce qui fait qu'à ce jour 18 allié 18 sur 30 ont déjà ratifié le protocole, parmi lesquels le Canada, le Royaume-Uni et nombre de pays européens dont l'Allemagne ou encore la Pologne aux États-Unis les 2 textes ont été approuvé par la Chambre des représentants et sont désormais soumis à l'examen du Sénat. ce matin, alors que je m'apprêtais à vous dire que 17 alliés avaient ratifié les protocoles, la Belgique vient d'achever son processus de ratification portant ce nombre, En France, le projet de loi autorisant la ratification de ces 2 protocoles d'adhésion examiné par le Conseil d'État le 12 juillet puis en conseil des ministres, le treize, il est désormais soumis à votre approbation. C'est ensuite notre responsabilité vis-à-vis de nos compétiteurs et rivaux stratégique jusqu'à leur adhésion effective, Stockholm et Helsinki ne seront pas formellement couverte par l'article 5 et pour être exposé à des actions de provocation de déstabilisation conduite par des pays hostiles à cet élargissement dont ils perçoivent bien qu'il réduira à terme leur marge de manoeuvre et leurs moyens de pression. Nous avons d'ailleurs fait part de notre disposition à apporter des mesures de réassurance pour cette période intermédiaire si la Finlande et la Suède, le souhaitent. Par ailleurs, et comme le président de la République l'a rappelé. Ces 2 pays bénéficie bien sûr de la clause d'assistance mutuelle de l'article 42 paragraphe 7 du traité sur l'Union européenne. Il en va enfin et peut-être surtout de notre responsabilité à l'égard de nos concitoyens dans la sécurité est notre priorité, nous pourrons assurer encore plus efficacement leur sécurité, en renforçant notre sécurité collective. La France participe pleinement depuis 2014 et plus encore depuis le 24 février dernier au renforcement de la posture de l'Alliance sur le flanc oriental, elle participe à la présence avancée de l'OTAN en Roumanie en tant que nation cadre et elle est présente également en Estonie, elle contribue aux opérations de police du ciel et de surveillance maritime dans l'espace considéré. Ainsi, comme l'a dit le président de la République, nous devons être au rendez-vous de l'histoire en menant à bien le processus de ratification de ces 2 protocole. Enfin je rappellerai que les dispositions de ces 2 textes sont pleinement compatibles avec d'une part, les engagements pris par la France dans le cadre des Nations-Unies, article 2, article 51 de la charte de l'autre, avec ses engagements dans le cadre de l'Union européenne, le traité sur l'Union européenne, article 42 7 que je mentionnais il y a quelques instants, renvoie effectivement aux engagements souscrits par les États membres dans le cadre de l'OTAN ainsi la ratification du protocole de ces 2 protocoles ne nécessitera-t-elle pas de modification du droit français, ou l'adoption de dispositions législatives ou réglementaires nouvelles. Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle le projet de loi visant à autoriser la ratification du protocole au traité de l'Atlantique nord sur l'accession de la République de Finlande et la ratification du protocole au traité de l'Atlantique nord sur l'accession du royaume de Suède aujourd'hui proposer à votre approbation, je vous remercie. rapporteur de la commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées. Monsieur le président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Qui aurait cru il y a seulement 6 mois que nous serions appelés à débattre de l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, si nous en avions besoin, voilà bien la preuve de la gravité de l'agression russe contre l'Ukraine et des conséquences innombrables que celle-ci entraîne en vérité vous l'avez dit madame la ministre, il s'agit bien d'un événement historique pour l'Europe, dont nous devons prendre conscience aujourd'hui mesures ont, en effet, la révolution mentale, le changement d'air que cet événement constitue, tant pour les Finlandais que pour les Suédois pour les premiers, les Finlandais, c'est un stigmate de la guerre froide qui soudain s'efface pourtant cette neutralité contrainte visait précisément à survivre à la menace russe le renoncement à une politique étrangère pleinement indépendante cette fameuse finlandisation ces sacrifices semble donc aujourd'hui insuffisant face à une Russie jugée plus menaçante qu'au pire moment du rideau de fer en 2020 20 % des Finlandais soutenait l'adhésion à l'OTAN, ils étaient 76 % en mai 2022, les autorités d'Helsinki avait tenté de conserver une approche équilibrée vis-à-vis de Moscou, tout ceci aura donc été balayée par l'agression russe loin d'aboutir à la finlandisation de l'Ukraine, l'aventure de monsieur Poutine a précipité l'OTAN Isa Sion, de la Finlande. Pour les Suédois, le séisme est sans doute encore plus violents et peut être plus profond en paix depuis 1814 ce pays peut se féliciter d'avoir échappé à toute invasion pendant de longs siècles et voici que veulent soudain en éclats un élément constitutif de l'identité nationale, fondée sur l'alliance étroite de la neutralité d'un soutien sans faille au multilatéralisme et d'une aide massive aux pays en voie de développement, la Suède avait lié depuis longtemps son destin à celui de la Finlande en matière de sécurité extérieure, il allait clair, il était clair que dans cette affaire de l'OTAN, la Suède allait emboîter le pas à la Finlande alors qu'apporte cette adhésion aux 2 pays et réciproquement qui porté la l'alliance et de ce fait, quel est son apport aussi pour nous, les Français l'assurance stratégique que représente l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord constitue évidemment la première motivation des 2 pays avec l'agression russe, la fameuse garantie de sécurité est sorti des manuels de droit international pour redevenir plus concret le plus précieux des remparts, pour la première fois depuis la fin de la guerre froide, plusieurs pays européens se sentent eux-mêmes directement menacés dans leur existence par la Russie. Les récentes déclarations américaines et de responsables de l'OTAN, selon lesquelles l'Alliance défendrai, je cite : chaque centimètre carré du territoire des pays membres n'ont fait que renforcer la valeur symbolique de cet article 5. Du point de vue de l'OTAN, il s'agit d'un succès considérable, on est passé en moins de 2 ans du constat d'une organisation en quasi mort cérébrale malmené par le président américain a une OTAN attractive et revivifier l'adhésion des 2 pays, dont la neutralité paraissait intangible marque ainsi une véritable résurrection. Sur le plan concret ensuite l'apport à notre sécurité collective n'est pas négligeable, bien au contraire, les armées de ces 2 pays sont complètement inter-opérable avec celle de l'OTAN, au-delà des mécanismes de coopération que vous avez rappelé : Madame la Ministre, ce lien a été forgé dans l'épreuve par les combats communs que nous avons menée dans les Balkans, en Afghanistan et en Irak, au terme de cette évolution qui s'est encore accélérée avec l'invasion de l'Ukraine, la Finlande et la Suède sont aujourd'hui et de loin, les 2 pays les plus proches de notre alliance il dispose aussi d'importantes capacités. Sans revenir longuement sur ce point qu'il suffise de rappeler que la Finlande touche déjà au fameux 2 % du produit intérieur brut consacré à la défense, seuil que la Suède a promis d'atteindre en 2028 la Suède, quant à elle, dispose d'une solide industrie militaire et a récemment réintroduit le service militaire obligatoire, tandis que la Finlande pour sa part peu modifier mobiliser jusqu'à 870000 réservistes. Toutefois, nous aurions tort de mesurer l'apport que constitue l'adhésion de ces 2 pays en nous contentant les d'additionner les uns aux autres, les milliards d'euros, les équipements ou les hommes tout comme nous aurions tort de croire que ces chiffres suffisent à assurer notre sécurité, j'y reviendrai dans une seconde, d'un côté, ces adhésions apporte en fait une profondeur stratégique nouvelle qui renforcera la posture de défense et de dissuasion du flanc oriental de l'OTAN ceci crée de nouveaux dilemme stratégique pour la Russie et permettra certainement une défense plus crédible des Pays Baltes, que nous avions visité récemment avec le président du Sénat, d'un autre côté, cet événement nous fait entrer dans une situation nouvelle, nous obligeant à redoubler de prudence, l'adhésion de la Finlande of à l'OTAN 1000 300 nouveaux kilomètres de frontière où il faudra à la fois contrer avec fermeté et discernement les inévitables provocations russes et éviter aussi tout risque d'escalade, le fait qu'Helsinki garde une tradition de bon voisinage avec la Russie et a un intérêt évident à garder la situation sous contrôle constitue de notre point de vue un atout indéniable, inversement, il faut souligner qu'aucune demande n'a été formulée en vue du déploiement de forces ou d'équipement de l'OTAN sur les territoires, suédois ou finlandais, ces 2 pays estimant eux-mêmes, être en mesure de se défendre. Je voudrais néanmoins aborder 2 points de vigilance très important pour nous même, Madame la Ministre, tout d'abord, et vous l'avez évoqué le chantage exercé par la Turquie, qui bloquait le processus d'adhésion n'a été surmonté qu', prix de la signature d'un mémorandum trilatéral et celui-ci peut interroger pour au moins 2 raisons : premièrement, la Finlande et la Suède se sont engagés en pas à empêcher les activités du PKK mais aussi du pays Grecs des des IPG qui sont nos alliés dans la coalition internationale contre Daech en Syrie, elle promet aussi de lever leur embargo sur la vente de certaines armes à la Turquie, ce qui peut poser problème. Autre point d'attention et de vigilance, Suède et Finlande se sont engagés à soutenir la participation de la Turquie aux initiatives de la PSD, c'est une telle participation ne va pourtant pas de soi, étant donné l'attitude actuelle de la Turquie envers la Grèce et Chypre, comme l'a souligné le rapport sur la boussole stratégique de nos collègues, Ronan Le Gleut : Hélène Conway au-delà d'un évident problème de compatibilité de valeur, il faut éviter que les bénéfices de ce genre de coopération ne s'avère déséquilibré au profit d'un pays qui, en l'occurrence ne respectent pas toujours les règles de l'OTAN, c'est le moins qu'on puisse dire, aussi est-il impératif de veiller à ce que le temps ne s'aligne pas sur un mémorandum qui par nature ne doit pouvoir engager ni l'Alliance ni les alliés vous en avait pris l'engagement, Madame la Ministre, et je vous en donne acte. 2ème point de vigilance cette double adhésion signifie certes un renforcement de l'OTAN, mais nous sommes en droit de nous poser la question, de quel temps nous parlons premièrement, l'entrée de la Suède et de la Finlande pourrait avoir des conséquences sur la politique de la dite de la porte ouverte, les candidats actuels sont l'Ukraine et on voit bien le problème que pose cette demande, la Géorgie et la Bosnie-Herzégovine ce sujet doit continuer à être abordée avec courage et lucidité chaque adhésion doit rester un processus individuelles liées à la mise à niveau de l'appareil de défense mais aussi à la situation politico-militaire de chaque candidat au-delà et c'est un second point d'attention, le sommet de Madrid a abouti à une révision du concept stratégique de l'OTAN, avec une mention inédite du fait que, je cite, les ambitions et les politiques coercitives de la Chine, remettent en cause nos intérêts notre sécurité et nos valeurs, en outre, le Japon, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande ont été pour la première fois, invité à assister à un sommet de l'OTAN. Nous pensons qu'à rebours de cette évolution vers une alliance globale, l'entrée dans l'OTAN de de pays membres de l'Union européenne doit au contraire être un levier pour renforcer la dimension proprement européenne de notre sécurité, la Suède et la Finlande, ce sont d'ailleurs engagés à renforcer la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN, ce dont nous nous félicitons remarquons tout de même que ces 2 pays sont déjà en tant qu'État membre de l'Union européenne, couverts par la garantie de sécurité de l'Arctique 42 7 du traité de l'Union européenne, autant dire que celle-ci a encore beaucoup à faire pour assurer sa crédibilité dans le même ordre d'idées, nous devons oeuvrer au sein de l'OTAN pour que ce nouvel essor profite au renforcement des capacités de défense propre aux pays européens. Sous ces réserves, la commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées vous propose donc de ratifier l'adhésion de l'à l'OTAN de la Suède, de la Finlande c'est de démocratie qui partage pleinement nos valeurs, vous venez de le rappeler 18 pays de l'OTAN et plus dans les heures qui viennent de précéder la Belgique, la Lituanie 18 pays de l'OTAN ont déjà ratifié les protocoles, nous avons encore quelques inquiétudes du côté de la Turquie, mais en attendant la fin du processus de ratification, il serait prudent de ce Sophie, il ne serait peu prudent de se fiait aux déclarations russes plus modéré qu'il y a 3 mois, sur ce sujet, c'est pourquoi nous nous félicitons que la France est proposé à la Suède et la Finlande, des mesures de réassurance que vous venez d'exposer en choisissant de rejoindre l'OTAN, la Suède et la Finlande ont fait un choix historique qui crée une communauté de destin encore plus étroite avec les autres pays européens au moment où nous devons opposer l'unité et la fermeté à une agression intolérable l'entrée au sein de l'Alliance, représente pour nous de la part de la Suède et de la Finlande et pour tous ceux qui soutiennent, du reste, l'Ukraine martyrisée un apport précieux tant en faveur de la paix que de notre propre sécurité, je vous remercie. Merci monsieur le président. Dans la suite de notre discussion générale, je vais donner la parole à Madame Nicole Duranton pour le Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants, vous avez la parole, ma chère collègue. Merci monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, président de la commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, lancée en février 2022 des demande formelle d'adhésion ont été Débo, déposé le 18 mai auprès du secrétaire général de l'OTAN : pas de pays de l'Union européenne, proche de l'Alliance, la Finlande et la Suède, c'est un moment historique, vous l'avez rappelé : Madame la Ministre, l'OTAN et la Suède, partage des valeurs communes, entretiennent un dialogue politique ouvert et régulier et mène une coopération pratique dans un large éventail de domaines la coopération a débuté en 1994 lorsque la Suède a rejoint le programme de Partenariat pour la paix, sa première contribution, une opération dirigée par l'OTAN remonte à 1995 lorsqu'elle a déployé un bataillon en Bosnie-Herzégovine au Kosovo, en Libye, en Afghanistan, la Suède s'est engagé aux côtés de l'OTAN de ce on, de ce côté, après 1947 la Finlande a pu rester une démocratie parlementaire et il n'a pas eu à intégrer le Pacte de Varsovie, en échange de ne pas rentrer dans l'OTAN et de refuser de bénéficier du plan Marshall, dans les années 1950 on a ainsi commencé à parler de finlandisation pour désigner la neutralisation d'un pays dans la sphère d'influence d'une grande puissance, toutefois, comme pour la Suède, la coopération a débuté en 1994 la Finlande a participé aux exercices de l'OTAN en Bosnie Herzégovine aux Balkans en Afghanistan, en Géorgie, en Albanie, en Moldavie et en Irak en 2017 à la créer dans sa capitale, le Centre d'excellence européen pour la lutte contre les menaces hybrides et signer l'accord-cadre Cyber défense l'OTAN a pleinement respecter la politique de non-alignement militaire de la Suède et de la Finlande, mais aujourd'hui, le temps de la finlandisation est dépassée, voire renverser, le fait que ces 2 pays neutre, demande à rejoindre l'OTAN témoigne de la gravité et du caractère inédit de la situation en Europe en Europe avec la guerre en Ukraine, en tant que nation, cela nous oblige les pays se sentant menacé, ne veulent plus isolés, se replier sur eux-mêmes, mais au contraire s'intégrer dans des structures plus grande, bien sûr, cela doit aussi se faire en cohérence avec la construction de l'Europe de la défense une OTAN élargie et forte peut tout à fait co-exister avec l'Europe de la défense, comme l'a rappelé hier, lors de son audition devant notre commission, notre ministre des armées, Sébastien Lecornu, c'est une volonté forte de notre président de la République, Emmanuel Macron, l'Europe s'étant toujours construite durant des périodes de crise, nous avons en face de nous, toutes les occasions d'avancer sur les questions de défense le quatre juillet à l'issue du sommet de Madrid, les pourparlers d'adhésion ont été menées à bien, au siège de l'organisation à Bruxelles, le lendemain, les alliés ont signé le protocole d'accession, qui doivent désormais être ratifiée par les 30 pays membres de l'OTAN, les 2 pays font partie des 6 partenaires une nouvelle opportunité, il participe au programme de transport aérien stratégique sac et ça lisse de science au service de la paix et de sécurité et la mise en application de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité comportant à sa création, 12 membres, l'OTAN s'est bien élargie 8 fois depuis 1949 pour accueillir 18 nouveaux membres expliquer en détails le processus d'adhésion peut paraître fastidieux mais il a pris moins de 2 ans pour la messe Adwan, du nord au vu de la situation, l'adhésion de ces 2 pays devraient vrai sans là vraiment être encore plus rapide, en effet, les différents critères à respecter, ne devrait pas poser de problème, le secrétaire général de l'OTAN s'est dit confiant sur les chances d'adhésion de la Finlande et de la Suède, mais les 2 pays sont tout de même ralenti dans leur demande d'adhésion par 2 facteurs bloquants, la Turquie, d'une part, la Russie, d'autre part, après leur avoir demandé de faire le nécessaire pour extrader les membres du Parti des travailleurs kurdes sur leur territoire en marge du sommet de Madrid fin juin, le président turc, Erdogan a accusé Stockholm et elle Nijinski d'auberges pour les terroristes du PKK, ce lundi 18 juillet il a à nouveau menacé de geler ses adhésions opérant un chantage à la veille du sommet tripartite avec la Russie et l'Iran à Téhéran le ministre des Affaires étrangères turc a été plutôt rassurant, en reconnaissant que la Finlande était très respectueux des inquiétudes du président Erdogan en fait la Turquie semble vouloir négocier la fin de l'embargo imposé sur ces drônes Vladimir Poutine affiche aussi son hostilité à cet élargissement de l'OTAN, dont il fustige les ambitions impérialistes au plan géopolitique, les Russes redoutent l'installation par l'OTAN d'un arc nucléaire à leurs frontières à ce jour, comme vous l'avez rappelé 18 membres ont déjà ratifié les protocoles inter-l'élargissement est conforme aux stipulations de l'article 10 du traité de l'Atlantique nord relatifs à la politique de la porte ouverte soutenue par la France au plan militaire, l'adhésion de la Finlande et de la Suède permettra ainsi à l'Alliance et donc à la France de bénéficier du potentiel de 280000 soldats 870000 réservistes finlandais et du poids de l'industrie de défense suédoise dans le cadre de leur adhésion à l'OTAN, la Finlande et la Suède s'engage à maintenir un niveau d'investissement militaire à hauteur de 2 % de leur PIB le bureau de la planification de l'OTAN a établi que la Finlande contribuerait à hauteur de 24 millions d'euros et la Suède, à hauteur de 50 millions d'euros au financement commun annuel de l'Alliance en conséquence la contribution de la France diminuera, une économie de plus de 5 virgule 4 millions d'euros pour le budget militaire est presque un 1000000 d'euros pour le budget civil selon l'estimation préalable faite par la représentation permanente française, bien entendu, le groupe RDPI est favorable à ce projet de loi autorisant la ratification de ces 2 protocole. Je vous remercie, merci, ma chère collègue il appelé le président Claude Malhuret pour le groupe, les indépendants, république et et territoires. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, président, mes chers collègues, l'histoire du 20ème siècle fut celle de la lutte à mort entre les démocraties et les totalitarismes parfois très près de la perdre, nous l'avons gagnée par 2 fois, la première à la chute du mur de l'Atlantique, la deuxième à la chute du mur de Berlin, nous avions cru cette victoire définitive le XXIe siècle nous apprend que nous ne trompe le 24 février 2022 ne marque une rupture que pour ceux qui ne l'avait pas encore compris l'invasion russe n'est qu'un épisode particulièrement sanguinaire du retour de cette lutte mortelle retour qui a commencé à Grozny et s'est poursuivie en ne sait, il en a Brazi en Transnistrie en Syrie, en Libye, aujourd'hui en Ukraine et en Afrique, demain en mer de Chine ne nous y trompons pas, ce n'est pas la Russie, qui va changer la donne avec son PIB égal à celui de l'Espagne, et malgré ses rodomontades nucléaires. C'est la Chine bientôt, première puissance mondiale qui est scrutée attentivement l'issue du conflit en Europe pour fixer sa stratégie face à Taïwan, hé face au monde démocratique. Les Américains le savent au moins depuis Obama les Européens auraient aimé conserver leurs illusions ils certains certains par mercantilisme, d'autre part, anti-américanisme, d'autres enfin, par lâcheté ou par naïveté que le bourreau le record devrait encore un instant. La sale guerre de Poutine, c'est atroce à dire nous a ouvert les yeux. Victime du piège de Thucydide, le tueur du Kremlin est allé trop loin, trop tôt il diviser l'Europe, il la cimente ridiculiser l'OTAN ils la retrouvent humilier les États-Unis ils ressuscitent Biden après le revers de Kaboul. Rallier les dictatures sous sa bannière, la Chine s'inquiète de cette erreur stratégique, la Turquie montre les dents, le Kazakhstan, refuse l'envoi de ces soldats, l'adhésion de la Finlande et la Suède à l'OTAN, est un symbole majeur de nos yeux, enfin ouvert, de même que les sanctions enfin efficace. L'aide militaire conséquente à l'Ukraine et la mobilisation unanime de toutes les démocraties, la prise de conscience a été là s'tardive, c'est toujours le point faible des démocraties croire en 2008 après la Géorgie qu'on pouvait continuer à être partenaire de la Russie, renoncer à répondre aux attaques chimiques dans la Ghouta en 2013 se borner à quelques sanctions lors de l'annexion de la Crimée en 2014 était la porte ouverte aux rêves de conquête du petit caïd de Saint-Petersbourg, devenu colonel du KGB cuit dictateur puis boucher ne recommençons pas ses erreurs à ceux qui espèrent le lâche soulagement d'une négociation par dessus la tête des Ukrainiens, il faut répondre que c'est aux Ukrainiens. De décider et qu'ils ont décidé de défendre jusqu'au bout leur liberté et la nôtre, à ceux qui craignent d'humilier, Poutine, il faut rappeler que pendant des décennies, ce sont les peuples d'Europe de l'Est qui ont été humiliés occupée, colonisée par l'Union soviétique, que c'est l'Ukraine qui est aujourd'hui humilié, massacré et détruite que toute solution autre que le retour de l'Ukraine dans ses frontières antérieures à 2014 serait sa défaite, celle des démocraties et du droit international, elle préfigurerait d'autres agressions d'autres conflits et d'autres défaite elle signifierait pour les alliés de l'Occident, la certitude d'autres abandons à Taïwan au Moyen-Orient, en Afrique ou ailleurs, et pour les pays qui hésite, elle serait la tentation irrésistible regardez déjà les votes à l'ONU de tomber du côté des dictatures, notre objectif doit être la défaite de Poutine, le 2ème, point faible des démocraties et celui du long terme face à une guerre qui affecte l'économie aggrave l'inflation augmente les dépenses d'énergies, il faudra tenir compte la mauvaise petite musique de la 5ème colonne des extrémistes de droite et de gauche poutinien hier munichois aujourd'hui renforcée par tous les trolls les bottes et les trash Médias viendra susurrer que la guerre coûte trop cher, que tout n'est pas noir ou blanc, que ce sont nous, les agresseurs, que ce n'est pas notre guerre alors que bien sûr elle est, n'en déplaise à ceux qui, ici ou à l'Assemblée s'apprête, honte à eux, a voté contre ce texte de ratification 3ème défi, la guerre a convaincu les Européens d'accepter enfin la bouteille la boussole stratégique proposée par Emmanuel Macron, qui jusqu'à présent prêcher dans le désert parviendrons-nous à ce réarmement et combien de temps mettront nous que j'ai un siècle d'affrontements des dictatures et des démocraties qui se rallume que les dictatures et les totalitarismes aujourd'hui la Russie demain la Chine portent en eux la guerre comme la nuée l'orage et qu'il faut choisir son camp, prétendre échapper à ce cadre géostratégique où il occupait une pollution édition de neutralité tout en comptant sur le parapluie américain serait une incompréhension des rapports de force l'Europe puissance ne se conçoit que dans une alliance toujours plus étroite avec les autres démocraties alliance qui assurent notre sécurité depuis 1945 et dans l'appartenance renforcé à l'institution qui incarne cette alliance depuis 1949 l'OTAN bienvenue à nos frères finlandais et suédois. Merci monsieur le président. Je vais donner la parole oh. Président Roger Karoutchi pour le groupe Les Républicains.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le président de la commission. Il y a quelques mois, Monsieur le Président, à votre demande, je recevais le président finlandais Sauli Niinisto. Et à ma grande surprise, pour être très franc, alors que nous avions des notes des rapports nous disant hou la la la Finlande ne veut pas bouger pour le moment, elle regarde comment s'arranger ou. Trouver en tout cas une voie de passage avec la Russie, le président finlandais me disait et j'ai immédiatement transmis au président du Sénat, en lien avec le Quai d'Orsay. Qu'il avait trouvé lui conservateur, président de la République depuis 2012 un accord avec sa première ministre social- démocrate Première ministre depuis 2019 pour dire nous voulons adhérer à l'OTAN, contrairement à tout ce qui se disait dans la classe politique finlandaises dans la classe politique suédoise depuis des années. Effectivement, je veux pas reprendre tout ce qui a été dit. Bien sûr, le groupe, les républicains je rassure tout le monde, je suis sûr que vous étiez inquiet va voter ce projet de loi oui je vous sentez nous Dire que c'est un énorme succès pour l'OTAN, oui, c'est un énorme succès d'avoir 2 états européens puissants, on l'a redit ayant vraiment de fortes armés, et il y a vraiment des consciences ayant un passé le président comme on l'a rappelé la Suède. Neutre depuis 2 siècles, depuis Bernadotte. La Finlande, malheureusement pour elle, Finlande disait contre son propre avis après la deuxième Guerre et après l'invasion soviétique de 1940 en Carélie. Mais c'est le résultat d'un échec quand même. C'est quand même le résultat du fait que l'agression russe en Ukraine. Ah provoqué en Europe de l'Est. Un mouvement sinon de terreur, du moins de très fortes inquiétudes. Si les pays baltes, si la Pologne ont adhéré, par le passé à l'OTAN, c'est bien pour participer pour être protégé par rapport aux géants russe voisin et aujourd'hui, la Finlande et la Suède se disent ça n'est plus possible de discuter, de négocier, de trouver des voies de passage avec la Russie, nous avons besoin du bouclier de l'OTAN, le président Cambon rappeler qu'il y a deux 3 ans non seulement on disait l'OTAN ce machin quasi mort on se demandait même s'il fallait pas y mettre un terme créer autre chose, on parlait beaucoup plus du Bouclier européen du modèle européen d'une armée européenne, de la capacité de l'Europe par elle-même et puis aujourd'hui. Le réalisme l'a emporté, et nous voilà dans toute l'Europe, bien content d'avoir les Américains. Et les États, comme la Finlande et la Suède s'empresse de revenir vers nous, alors que, il pourrait dire bah déjà dans l'Union européenne avec l'article 42 7 nous avions cette solidarité mais nous préférons avoir en plus l'article 5 du parc de l'Atlantique nord, il y a donc effectivement un 1er résultat à l'agression sauvage de Poutine en Ukraine, c'est le fait qu'il a ressuscité la volonté européenne de participer à l'OTAN et qu'il a ressuscité en France, le fait que toutes les opinions publiques qui, très divisés sur l'OTAN, finalement font bloc, en se disant : quand on voit ce qui se passe en Ukraine et ben, on se retrouve plutôt en accord avec le fait que naturellement nous pouvons participer tous ensemble à cette force qu'autant alors on l'a dit et je ne vais pas être très long, puisque les choses sont claires pour nous. C'est une force supplémentaire. La Finlande à 1300 kilomètres de frontières et elle le sait, elle a durement payé dans le passé avec la Russie, Poutine est un peu imprévisible, il faut quand même dire les choses parce que, en France ou ailleurs, madame la Ministre, au début de cette année, on nous affirmait que, au final, il y aurait pas d'invasion russe de l'Ukraine puis l'invasion et la et à partir du moment où l'invasion et là les gens réagissent avec émotion avec toutes les tensions que ça veut dire et nous sommes évidemment partie prenante. On l'a dit, cette adhésion entraîne un nouveau chantage du maître d'Ankara chantage sur le PKK chantage sur les mouvements avec lesquels nous avons, nous avions désaccord dans la lutte contre Daech jusqu'où l'OTAN jusqu'où les pays membres de l'OTAN doivent aller pour satisfaire la Turquie et à empêcher la Turquie de bloquer l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, c'est un vrai enjeu, j'ose espérer, Madame la Ministre, que naturellement vous l'avez dit, ce n'était pas un engagement de l'ensemble de l'Europe et de l'ensemble de l'OTAN, mais seulement de de la de la Suède, mais enfin quelle est l'étape suivante, pour le moment, la Turquie n'a pas donné d'accord sur l'adhésion est ce que nous n'allons pas avoir dans les derniers jours de nouvelles demandes de nouveau chantage, que le gouvernement turc avait à nouveau à 2 voix, d'un côté les durs, qui disait : on n'a pas obtenu assez, il faut obtenir plus pour accepter l'adhésion de l'autre, les diplomates qui eux évidemment essayer d'enrober tout ça, mais enfin, ça veut dire quand même que c'est vrai, nous sommes contents que la Finlande et la Suède adhère à l'OTAN, mais c'est pas facile tous les jours, de gérer l'OTAN avec la Turquie. Il y a donc un problème permanent sur la vie sur l'avenir de l'OTAN et puis les orateurs précédents l'ont dit, moi, je ne sais pas ce qui va se passer avec la Chine, mais enfin, hier, je voyais des. Non pas des délibérations, mais les annonces faites par des organismes chinois certes pas le gouvernement mais par des organismes chinois qui commençait à dire Taïwan, ça n'est plus qu'une question de semaines, sous-entendu : bah, l'affaire ukrainienne finalement semble dire que on peut peut être avancé alors bien sûr, les États-Unis sont là, la flotte américaine et la la protection de Taïwan et là, mais là encore, madame la Ministre et je j'arrêterai par là. Dans le son. Poutine non seulement a ressuscité Bagdad. Mais il a ressuscité la volonté d'hégémonie américaine parce que voilà : les États-Unis champions en Europe champions en Ukraine avec une industrie militaire capable de fournir à tous les États qui, dans l'inquiétude augmentent leurs crédits augmentent leurs Budgets militaires et qui donc vont passer des commandes et l'industrie militaire américaine va très bien s'emporter. Et puis voilà, les États-Unis qui, en Asie, nous disent oui français : vous avez toujours dit que vous aviez un modèle indo-Pacifique et que vous avez la Nouvelle-Calédonie que vous vouliez négocier avec l'Australie, plus ou moins bien que vous vouliez négocier avec les uns les autres est-ce que vous n'allez pas être obligé de vous aligner sur la position américaine par rapport à la Chine, parce que dans l'ensemble mondial bah tout est lié, Poutine se rapproche de la Chine, donc les États-Unis soutiennent, Taïwan, les États-Unis soutiennent l'Europe, les États-Unis, vous pousse à rentrer à participer à l'OTAN attention madame la Ministre, oui nous sommes évidemment tous d'accord en France pour soutenir l'Ukraine oui, évidemment, nous sommes tous d'accord pour condamner la Russie oui, évidemment, nous sommes tous d'accord, peut-être pas tous d'ailleurs pour dire que l'adhésion de la Finlande et la Suède, c'est une bonne idée, c'est pour protéger des nations européennes qui peuvent en avoir besoin et qui ont intérêt à avoir un bouclier, mais en même temps, Madame la Ministre, moi j'ai entendu le président de la République, parler de la boussole stratégique européenne de la souveraineté de de l'Europe, attention à ce que la crainte, la peur, l'invasion de l'Ukraine, la crainte de ce qui peut se passer à Taïwan ne fasse pas finalement des États-Unis, le seul. Pays capable de fédérer par rapport à la crainte par rapport aux par rapport aux dictatures et par rapport au fait de défendre les démocraties, l'Europe doit exister davantage l'Europe doit imposer dans certains cas, sa vision, moi je pense que vous l'avez dit, d'ailleurs, Madame la Ministre, dans plusieurs déclarations, la boussole stratégique, la force de l'Europe doit se manifester, oui à l'adhésion de la Suède et la Finlande mais oui aussi à ce que l'Europe conserve sa puissance, sa force et ne soit pas uniquement à la traîne des autres. Et donner la parole au président Guillaume Gontard pour le groupe écologiste solidarité et territoires.

nous examinons, dans des conditions d'une extrême d'une extraordinaire urgence justifié par un bouleversement géopolitique tout aussi extraordinaire, la demande d'adhésion de la Suède et la Finlande à l'Organisation du traité de l'Atlantique nord, cela a été dit et redit, jamais au regard de la neutralité historique imposée ou pas de ces 2 pays, nous n'aurions imaginé la tenue d'un tel débat il y a encore quelques mois, cette volonté de la Suède et de la Finlande, de rejoindre l'Alliance Atlantique, mettant fin à des siècles pour l'une des décennies pour l'autre de neutralité militaire illustre avec force le bouleversement extraordinaire de l'ordre mondial. Et des équilibres géopolitiques européen provoquée par l'invasion la l'invasion pardon russe de l'Ukraine, 31 ans après la chute de l'URL, l'URSS, l'OTAN a brusquement et malheureusement retrouvé sa raison d'être. Ce retour de la puissance américaine aux Affaires européennes, quelque peu délaissé depuis le début de la présidence Obama est également hein, c'est nouveau, qui n'est pas sans interroger elle illustre en tout cas la faiblesse réelle ou ressentie de l'Union européenne à assurer sa sécurité collective le souhait de la Finlande et la Suède, de rejoindre l'OTAN témoigne de la confiance toute relative que ceux des pays porte à l'article 42 du traité de l'Union européenne qui garantit l'entraide militaire mutuelle entre ses membres, cela interroge sur l'efficacité de l'action diplomatique de la France ou plus accessoirement sur l'influence politique des écologistes pour oeuvrer en faveur d'une défense européenne collective, je ne ferai pas mystère des positions historiques de ma famille politique qui a toujours milité pour le développement d'une défense européenne à même de renforcer l'autonomie diplomatique et stratégique du continent vis-à-vis du partenaire états-uniens. Je n'aurais pas imaginé ça a été dit, me retrouver un jour dans la position de plaider avec force pour un élargissement de l'OTAN, mais comment pourrait-il en être autrement, comment, alors que la Russie agresse l'Ukraine et menace la Suède et la Finlande ne pas répondre favorablement à leur demande, souveraine démocratiquement, concertés d'adhésion à l'Alliance, comment pourrions-nous envoyer à la Russie et au monde, un tel message de désunion et de faiblesse, il n'est pas acceptable de briser la solidarité des pays occidentaux, qui est la seule voie possible pour permettre à l'Ukraine de sortir victorieuse de ce conflit et ainsi rétablir la paix sur le continent. En cohérence avec le soutien sans faille à apporter au peuple ukrainien par les écologistes européens, c'est tout naturellement que nous soutiendrons la demande de la Suède et de la Finlande rejoint la sécurité collective qu'apporte l'OTAN aux pays européens, c'est le prix de la défense de la démocratie, de la liberté et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes faut aux frontières orientale du continent, comme l'a excellemment montré le rapport de la commission commis dans la plus grande urgence, qu'il me soit permis d'ailleurs de saluer ici le professionnalisme professionnalisme de notre administration, il n'y a aucune difficulté juridique, économique ou militaire à intégrer ces 2 pays qui remplissent tous les critères fixés par le traité fondateur de l'Alliance fidèle donc à nos positions historiques, je formule le voeu, et je crois sincèrement que l'intégration de nouveaux pays jusque-là profondément isolé à l'effort collectif européen est une Pierre supplémentaire à la construction d'une défense collective, elle s'inscrit d'ailleurs dans une épisode dans un épisode historique de réarmement et de renforcement des capacités de défense des pays de l'Union européenne, au pire, au 1er rang desquels l'Allemagne, en effet, c'est le paradoxe de la période, le regain d'intérêt de l'OTAN n'est peut-être que conjoncturel en tout cas le renforcement de l'alliance ne peut passer que par le renforcement des capacités propres des pays européens, objectif compatible avec celui d'une Europe de la défense, c'est l'objectif de la France, rappeler avec force lors du sommet de l'Alliance des 28 29 et 30 juin dernier que de renforcer la relation Union européenne autant et d'insister sur le renforcement du pilier européen au sein de l'Alliance, les écologistes soutiennent cette position française je conclurai donc mon propos par 2 préoccupations qui ont été rappelés par plusieurs. De mes prédécesseurs, le protocole d'adhésion ne le prévoit pas mais rappelons clairement cet élargissement qui comportera désormais 1250 kilomètres de frontière supplémentaire avec, sur la Russie ne saurait se traduire par le déploiement de forces de l'Alliance en Finlande et en Suède, la situation est suffisamment conflictuelles avec le belligérants russe pour ne pas ajouter inutilement de l'huile sur le feu, un dernier mot pour dénoncer le chantage inacceptable de la Turquie, qui demande à la Suède, l'extradition de 33 membres du PKK en échange de la ratification du présent traité nous faisons confiance au royaume de Suède au regard des positions déjà exprimées pour ne pas céder et en aucun cas céder au chantage, les Kurdes qui n'ont de cesse de nous protéger contre la menace du terrorisme islamiste, non pas à être les victimes collatérales de la guerre en Europe, merci. La parole est maintenant notre président, Pierre Laurent, pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Vous avez la parole monsieur le président. Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, nous engageons donc au pas de charge la discussion pour valider l'adhésion de la République de Finlande et du royaume de Suède à l'OTAN, le gouvernement a ajouté ce projet de loi à l'ordre du jour, le 16 juillet nous votons 5 jours plus tard, une procédure exceptionnelle expéditive dans un hémicycle peu garni pour une décision pourtant de porter majeures dans le contexte de guerre actuelle, ce n'est ni sérieux ni responsable, on nous demande de ratifier les adhésions de ces 2 pays déjà validé au nom de la France au sommet de l'OTAN le 28 juin sans aucun débat approfondi une évaluation parlementaire préalables sur la nouvelle doctrine révisé de l'OTAN à Madrid dans laquelle ces adhésions s'inscrivent de fait l'agression inacceptable de la Russie contre l'Ukraine et les crimes qu'elle entraîne depuis ont ouvert une nouvelle page dangereuse de l'histoire des relations internationales, parmi toutes ces conséquences dangereuses pour la paix du monde, elle provoque aujourd'hui le basculement historique de de pays ancré de longue date dans la neutralité vers le ralliement à une logique du bloc militaire atlantiste au moment même où celui-ci durcit sa logique agressive qui peut sérieusement y voir une bonne nouvelle pour la sécurité internationale. Comme membre de l'Union européenne, la Suède et la Finlande pouvait déjà faire appel aux clause d'assistance mutuelle des traités européens, leurs armées sont déjà interopérables avec celles de l'OTAN dans le cadre du partenariat euro- Atlantique plus que sécuritaire, la décision est donc politique et géostratégique, ce qui change, c'est leur intégration systémique dans un dispositif sous commandement otaniens, autrement dit sous commandement américain seront-ils mieux protégés, où sommes-nous en train de les transformer en première ligne de front potentiels entre sans l'OTAN et la Russie, donnant ainsi, comme il est dit de la profondeur stratégique à l'OTAN nous prétendons les protéger quand nous les exposons encore plus au danger d'autant que si l'installation de bases militaires sur leur sol est, aujourd'hui, elle pourrait advenir à tout moment à l'avenir ces questions mériteraient un débat approfondi car la politique d'extension de l'OTAN, loin d'être un facteur de paix, a déjà par 2 fois au moins directement contre contrecarrer l'opportunité de travailler à de nouvelles architectures de sécurité collective paneuropéenne après la chute du mur de Berlin et la fin du Pacte de Varsovie ou un autre chemin était alors possible et après la première guerre de 2014 quand les accords de Minsk ont ouvert une voie laissée en jachère aujourd'hui l'escalade continue du côté de la Russie et du côté de l'OTAN, jusqu'où, sous impulsion américaine la doctrine révisé par l'OTAN à Madrid assume un tournant particulièrement inquiétant, elle va pousser un surarmement massif dans toute l'Europe et renforcer la logique mondiale d'affrontement de blocs militaires quand les grands défis de sécurité mondiale sont alimentaire, énergétique, climatique sociaux des centaines de milliards d'euros supplémentaires vont être engloutis par les pays européens membres de l'OTAN, dans les dépenses militaires, alors que l'OTAN représente déjà plus de la moitié des dépenses d'armement du monde, 3 fois plus que la Russie et la Chine réunit ses dépenses profiteront pour l'eau, pour au moins les 2 tiers aux industries d'armement américaines élargir l'OTAN accroître encore la tutelle américaine sur l'Europe et perdre un peu plus la bataille de l'eau, l'autonomie stratégique européenne la doctrine stratégique de l'OTAN en dose d'ailleurs pour la première fois l'élargissement de ses objectifs à la Chine, progressant vers l'objectif américain d'une alliance militaire à vocation mondiale, tourné à la fois vers l'Europe, l'Asie et l'Afrique, enfin, comment ne pas dire notre indignation devant le mémorandum signé entre le dictateur et maître chanteur Redjep Tayyip Erdogan pour marchander son appui à cette double adhésion la manière dont l'alliance et notre gouvernement minimise ce mémorandum de la honte et scandaleuse, les faits sont là nous trop con, contre le feu Vert turc l'extradition de démocrates kurdes pour les livrer à Erdogan qui, après une parodie de justice les laissera pourrir dans les prisons turques est ainsi que nous remercions les Kurdes qui ont versé leur sang pour combattre Daech l'hypocrisie qui consiste à prétendre que ce même Random trilatéral n'engage ni l'Alliance, ni la France ne fait qu'ajouter à l'indécence de la validation de facto par la France de ce deal indigne avec un dirigeant turc qui se tenait sommet il y a 2 jours avec Poutine et l'Iranien Ebrahim Raïssi à propos de la Turquie, je vous repose la question, madame la ministre, à laquelle vous ne m'avez pas répondu en commission, tout le monde craint une nouvelle offensive contre les forces kurdes dans le Nord-Est de la Syrie des frappes ciblées ont déjà eu lieu ces derniers jours qu'attend la France pour réagir et dénoncé ce nouveau coup de force, le chantage otaniens est-il le prix de ce silence coupable pour toutes ces raisons, vous le comprendrez, nous allons nous opposer à ce nouvel élargissement de l'OTAN, tout semble se résumer dans notre esprit à préparer la guerre nous attendons pour notre part, l'ouverture de débat urgent sur la relance de voies nouvelles vers la paix, celle de l'indépendance et de l'autonomie stratégique, celle de nouvelles architectures de sécurité collective incluant la solution politique des conflits intra-européens, toujours non résolu, je pense à Chypre et aux Balkans, celle de la relance du désarmement multilatéral ces voies nouvelles pour une sécurité humaine globale sont attendus dans le monde entier par une majorité de pays du monde, qui refuse l'alignement dans la logique des blocs pour son avenir, Madame la Ministre, la France devraient écouter la voix du monde, pas seulement celle du Bloc atlantiste, je vous remercie. Merci monsieur le président. La parole est à notre collègue Philippe Folliot pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président, rapporteur de la commission mes chères et chers collègues, il est des moments où les peuples ont rendez-vous avec l'histoire avec leur histoire. Il est des moments particulièrement important pour les démocraties avec la nécessité de prendre en compte leur défense. Ce qui s'est passé au mois de février dernier avec cette scandaleuse agression de l'Ukraine par la Russie ou pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, sur le continent européen, un État agressé n'en traitant a eu un certains nombres de conséquences. Parmi ces conséquences, c'est celle d'une prise de conscience de la fragilité de la sécurité collective telle que nous l'avions imaginé telle que nous la pension, j'allais dire quasiment éternel sur le continent européen. Et ceci a entraîné le fait pour nos amis finlandais et suédois, cette prise de conscience et cette volonté de rejoindre l'OTAN, somme toute, monsieur Poutine malgré lui a sorti l'alliance de ce n'encéphalogramme plat pour lui redonner une forme d'attractivité. Et nous ne pouvons que nous en réjouir. Au regard de cette situation, bien entendu, le groupe Union centriste apportera son soutien à ce projet de ratification. Il est pourtant important et est essentiel même de rappeler un certain nombre de points et je vais pas revenir sur ce qu'on dit, nombre de nos collègues, au regard de l'intérêt qu'il y aura pour l'alliance de cette double adhésion sur les conséquences au travers du fait de l'importance, j'allais dire de l'outil militaro-industriel suédois de, de, de l'importance de de la Finlande, notamment au travers de ses forces propres propres et réservistes 670000 réservistes et est un chiffre quand même, et qui nous fait envie à à certains égards, mais au-delà de de l'ensemble de ses de ses je crois que nous pouvons en profiter pour réfléchir ensemble et se poser un certain nombre de questions : la première, hein, c'est de constater que, somme toute, nos amis et partenaires et alliés suédois et finlandais ont préféré la protection de l'article 5 de l'OTAN à celle de l'article 42 alinéa 7 du traité de l'Union européenne, ceci doit nous interpeller parce que, au regard de tout ce que nous avons dit depuis bien longtemps sur les notions de sécurité collective à l'échelle européenne et de l'autonomie d'une forme de défense européenne, cette malheureusement à certains égards un cruel constat d'échec par rapport à cela. Bien entendu, nous devons aussi continué à porter nos éléments de réflexion parce que un des éléments de spécificité de l'OTAN, créée le 4 avril 1949 à Washington, c'est quelque temps après la création de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, c'est-à-dire que, pour la première fois dans une organisation internationale militaire à côté se trouve une organisation démocratique avec les parlementaires de tous les pays membres et d'un certain nombres de pays partenaires et du reste, nos collègues parlementaires suédois et finlandais nous accompagne et et son auprès de nous, dans le cadre des éléments de réflexion au sein de cette assemblée parlementaire de l'OTAN, donc j'ai l'honneur d'être d'être mais nous devons aussi profiter de l'occasion pour réfléchir sur effectivement les enjeux relatives aux aux nouvelles candidatures qu'il y a au sein de l'OTAN, il y en a trois à ce jour formellement formaliser la Bosnie, la Géorgie et l'Ukraine, qui est dans une situation un peu particulière, il est clair que nous devons Sandy, chacun de ces à leur agissement en fonction des éléments d'opportunités et des difficultés et des problématiques que cela pourrait poser ensuite, nous devons aussi en profiter pour dire que si l'alliance aujourd'hui est obnubilée par ce conflit de relative à à l'Ukraine et à la Russie, nous ne devons pas pour autant oublié les autres défis stratégiques qui concernent à l'alliance, il y a celui de la question qui est toujours pas résolu des difficultés sur les Balkans occidentaux et nous y avons réfléchi à de multiples reprises au sein de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, mais aussi la situation du Sahel qui est un élément d'interrogation et pour lequel, du reste, c'est une des spécificités de la délégation française, chaque fois, de rappeler ces enjeux relatifs au Sahel au Moyen-Orient, en gros, pour reprendre une expression chère au président quand bon le flanc sud qui ne doit pas être oubliée par rapport par rapport à cela, mais si ces questions sont des questions éminemment importante, nous devons pas non plus être dupe et être naïf au regard d'un certain nombre de considérations concernant l'OTAN, c'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui au travers de la Turquie au travers qui nous interpelle, par rapport au au processus de ratification et et et aux éléments qu'il pourrait y avoir et aux mauvaises surprises que nous pourrions avoir, in fine, et dans ce cadre-là, parce que la séparation des pouvoirs que nous revendiquons dans notre démocratie, ici en France, est aussi vrai en Turquie et on pourrait craindre un certains nombres de jeux de rôles entre guillemets entre exécutif et législatif, ne faisons pas de procès d'intention, par rapport à cela mais, pour autant, soyons lucides, mais nous avons aussi un certain nombre d'autres points et d'autres enjeux relative au fait que les Américains ont repris la main et que dans ce cadre-là, ne nous y trompons pas, leur objectif est de favoriser les exportations sur étagère d'armement notamment dans nombre de pays européens et ceci donc nous interpelle sur la stratégie européenne en matière d'industrie de défense et la nécessité de structurer celle-ci et la problématique du lien entre l'Union européenne et l'OTAN par rapport à ces enjeux, d'autres, d'autres questions qui seront un jour ou l'autre des questions très prégnante, il y a la volonté de la part des Américains aussi d'élargir, j'allais dire le le cadre de l'OTAN et et se poser la question de savoir si, somme toute, celle-ci ne devrait pas aller vers des enjeux au niveau du Pacifique, je crois que nous saurons tous d'accord pour dire que l'OTAN est une organisation régionale relatives à l'Atlantique nord, relatives à l'Europe, et relative à cette partie du monde et qu'elle ne saurait en aucun cas être entraîné dans des enjeux dans des schémas qui dépasserait le strict continent européen, je crois que c'est un élément important parce que n'oublions pas que, il y a quelques quelques mois l'article que 4 de notre organisation, donc de l'OTAN a été sciemment violé par 2 États membres donc les États-Unis et la Grande-Bretagne pour ne pas les nommer au niveau donc de l'opération aux cuisses, sans parler du rôle trouble d'un allié historique que nous avons, qui est l'Australie et que donc dans ce cadre-là, il est important et essentiel aussi donc d'avoir un mémoire l'ensemble de ces enjeux, donc pour toutes, toutes ces raisons, c'est avec lucidité, mais aussi avec enthousiasme parce que chaque fois que la famille des démocraties à l'échelle européenne ben se consolide, pour travailler donc sur ces enjeux de sécurité collective, c'est une bonne nouvelle, hé bien notre notre votera favorablement à la ratification, donc de ce traité d'adhésion de ces pays et donc nous leur souhaitons bienvenue au sein de cette famille de l'OTAN tous ensemble, nous essaierons de faire ce qu'il faut pour relever les défis de cette organisation et les défis de sécurité collective donc, finalement, nous nous rendons compte qu'ils sont éminemment merci. Merci. La parole est de notre collègue André Guillaume. Pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Je ne connais Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président, rapporteur de la commission, mes chers collègues, tout a été dit sur les bénéfices incontestables d'une adhésion de la Suède, de la Finlande au traité de l'Atlantique nord, tout d'abord, selon le vieil adage l'union fait la force, un passant de 30 à 32 membres l'OTAN au moins trois fort logiquement ses capacités militaires. Les 2 pays disposent en effet de moyens significatifs, notamment côté finlandais et ça a été dit, les ressources humaines très conséquente côté suédois, on observe de Stockholm que dispose une industrie de défense compétitive sur le plan stratégique, clairement, avec la fin d'une neutralité historiquement bien chez ces 2 pays, le flanc oriental de défense du continent européen trouverez se j'ajouterais, comme cela a été dit par le président et Madame Madame la Ministre, que les partenariats de défense déjà existant entre l'OTAN et ces 2 pays, règle la question de l'inter-opérabilité, cette perspective est donc très positive pour la sécurité collective du continent européen, ainsi que pour l'approfondissement du concept euro-Atlantique dans ces conditions, mon groupe est favorable au projet de loi qui nous est soumis, aujourd'hui j'ai vous tout de même quelques inquiétudes, les inquiétudes que nous sommes nombreux à partager au regard des dérives de Vladimir Poutine, la Finlande et la Suède souhaite adhérer sans délai à l'OTAN, j'en profite, Madame la Ministre, pour saluer la promptitude de la France et celle de nos nombreux alliés qui se sont vite engagés dans le processus de ratification, le souci, on le sait, ça a été dit vient du côté turc, sommes-nous certains qu'Ankara ratifiera rapidement, des accords ont été conclus sont-ils solide et compatibles avec les engagements du à une partie des Kurdes, qui lutte contre Daech ensuite si la reconnaissance de l'OTAN fin fin juin à Madrid est une bonne chose sur le plan capacitaire, elle signifie aussi une forme d'août nisation de l'Europe dans ce contexte comme sincère, la boussole stratégique porté par l'Union européenne et que la France a défendu activement pendant sa présidence européenne, ça fait en concurrence à l'OTAN et, dans une parfaite complémentarité, l'Union européenne doit conserver une certaine autonomie, un terme de décisions stratégiques la guerre en Ukraine se déroule à ses frontières et les défis qu'elle doit régler au sud au Sahel, en particulier la concerne aussi directement par le impact interne obligatoire migratoire et sécuritaire, en outre, le renforcement du pilier européen au sein de l'OTAN ne doit pas conduire à alimenter seulement, l'industrie de défense américaine au détriment de l'industrie européenne aujourd'hui 60 % des achats militaires européens proviennent des états des je félicite, je me félicite que Bruxelles condition de le projet d'acquisition conjointe de matériel à hauteur de 500 millions d'euros au principe d'achat des producteurs basés en Europe et sous contrôle européen, la fin de l'ère des restrictions budgétaires en matière de défense qu'implique le retour de l'OTAN me conduit, pour conclure, a déploré un paradoxe, à un moment où l'humanité court de graves dangers climatiques et jusqu'à envisager sa disparition que nous avons ici une grande priorité devant nous, nous voilà amenés à augmenter nos dépenses militaires pour faire face aux régimes autoritaires qui cherche à affaiblir nos démocraties, ce qui m'apparaît comme une ineptie le défi environnemental exige des moyens colossaux, faute de quoi, ce ne sera pas que la guerre mais une terre meurtri qui signera notre perte malgré ces réserves, la guerre en Ukraine et la posture martiale de la Russie nous oblige à considérer l'élargissement du pilier européen de l'OTAN comme incontournable, mon groupe le Rassemblement démocratique et social européen, il est donc favorable et votera donc dans ce sens, je vous remercie. cher collègue donner. La parole monsieur Stéphane Ravier pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste de d'aucun groupe. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, il nous est demandé de ratifier l'accession de la République de Finlande et du royaume de Suède à l'Organisation du traité de l'Atlantique nord, la portant à 32 pays en 2022, une question se pose, dans quel but aujourd'hui au sein de cette organisation, l'absence d'unité de vue les conditions d'une impuissance collective, cela revient à réduire l'autonomie des états souverains européens en les soumettant aux exigences américaines dont les intérêts sont souvent divergents des nôtres pendant ce temps, la Russie tente de faire revenir dans son giron les anciennes provinces soviétique, la Chine fourbit ses armes contre Taïwan et la Turquie, pourtant membre de l'OTAN entretient le mythe de l'Empire ottoman, en soutenant l'invasion de la province arménienne indépendante d'Artsakh par l'Azerbaïdjan en occupant militairement une partie de Chypre et en adoptant une attitude belliqueuse envers la Grèce en mer Égée ces impérialisme poursuivent leur propres enterrer leurs propres destinée et il en va de même pour le Bloc nord-américains qui trouvent dans la guerre actuelle en Europe l'occasion parfaite pour ne pas dire l'opportunité d'élargir son emprise et de souder les États liés au sein de l'OTAN contre l'ennemi russe, résultat les embargos à l'égard de la Russie, favorise les exportations des produits américains et notamment dans le domaine énergétique, et nous sommes condamnés, nous nous auto-condamnons aux pénuries et à l'inflation, élargir l'OTAN, c'est réduire le monde au conflit entre 2 blocs anéantir la 3ème voie et des tampons entre les États-Unis et la Russie, avec un tel scénario : le risque de conflit mondial est nous rendons potentiellement belliqueux de pays culturellement, habitués à la neutralité en les forçant à intégrer le principe de défense collective, tout en rendant progressivement inatteignable l'unanimité nécessaire à l'action, le président de la République en 2019 l'avait pourtant affirmé, l'OTAN est en état de mort cérébrale, à quoi bon dès lors avoir intégré encore l'année dernière la Macédoine du Nord et intégrer la Finlande et la Suède aujourd'hui issu de la guerre froide dessert nos intérêts souverains, nous a conduit à baisser nos Budgets de défense au point de devoir nous en remettre de nous soumettre au protectorat américain, l'autre l'OTAN sous l'égide des Américains, c'est l'échec en Afghanistan et nos 90 valeureux soldats morts pour l'honneur, ce sont les bombardements de civils et la guerre fratricide en Serbie, c'est la déloyauté d'alliés comme les États-Unis, qui mettent sur écoute nos dirigeants ou comme la Turquie qui brandit régulièrement la menace migratoire et agressent nos bâtiments de marine en Méditerranée la pragmatique Allemagne ne croient plus dans le mythe otaniens, elle a pris le tournant du réarmement 100 milliards pour moderniser son armée et possède désormais un budget annuel de défense fois supérieur au nôtre, dans le conflit russo-ukrainien, la vocation de la France devrait être pour retrouver sa tradition de non-alignement diplomatique de dialoguer pour préserver l'espoir de paix dans cet esprit, je m'opposerai à l'élargissement de l'OTAN, comme je me refuse d'ouvrir la porte à l'entrée de l'Ukraine, en son sein, je vous invite donc, mes chers collègues en faire de même afin de retrouver notre indépendance, notre efficacité et notre stabilité. Merci qui la parole est à notre collègue Jean-Marc Todeschini pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Paul, mon cher collègue. Merci monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, chers collègues. La succession des événements récents nous démontrent qu'en matière de géopolitique, il y a pas de certitude absolue, c'est l'histoire et la géographie peuvent venir éclairer les analyses des gouvernants, les nécessités immédiates emporte souvent les décisions ici le rôle de notre chambre est essentiel : nos débats doivent permettre d'éclairer celles et ceux qui nous succéderont auront un jour à prendre leur part sur la la conduite de notre pays en ce sens, nous devons toujours nous efforcer d'aller plus loin dans nos échanges que ne le laisserait penser le simple résumé de notre vote, cela est d'autant plus important sur un sujet comme celui qui se présente aujourd'hui en séance l'adhésion de la Finlande, de la Suède à l'étang ne nous cachons pas derrière de faux semblants, les nécessités de l'actualité, font que le vote de ce jour laisse peu de place au doute, naturellement, nous souhaitons que la ratification définitive de ce protocole d'adhésion ne soit pas à la fin, l'occasion d'un chantage à l'abandon de nos alliés kurdes dans un contexte où le dirigeant de la République fédérale de Russie s'est mué en assaillant aux portes de l'Union européenne, attaquant l'Ukraine un pays souverain à nos frontières, il est évident que les autres pays géographiquement proches vont rechercher toutes les voix leur permettant d'assurer la protection de leur population et l'intégrité de leur territoire, la première observation, c'est que ce sont bien les gouvernements de la Suède et de la Finlande, qui demandent à entrer dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord, en cela, les gouvernements de ces 2 pays s'adapte à une nouvelle réalité géopolitique soudainement suite à l'agression de la Russie, ils répondent aussi à une demande interne de leurs citoyens jusqu'alors historiquement attachée à la neutralité et on en a nuance singulièrement vis-à-vis de leur voisin russe, pour dire les choses clairement, cette demande n'est pas contrainte par les États-Unis, ou un autre État occidental. Elle ne répond pas non plus à une stratégie d'encerclement de la Russie, porté par les pays occidentaux, que ce soit au sein de l'OTAN ou de l'Union européenne mais bel et bien par la mutation d'un état voisin, a un potentiel agresseur ayant lui-même démontrer qu'il ne se contentait plus de mots mais était capable de passer à l'acte à tout, on est sur simple décision de son président absolu Poutine en ce sens, aucun autre débat état, encore moins un État européen ne saurait abandonner la Suède et la Finlande à leur sort, la solidarité ne peut être autrement quand hier et assumer cette nécessaire solidarité ne doit pas nous empêcher d'observer et de questionner le sujet de l'adhésion à l'OTAN en 2022, de 2 membres de l'Union européenne depuis 1995 en effet, dans notre analyse, nous ne pouvons pas masquer le fait que cette demande vient mettre en lumière une réelle faiblesse de l'Union européenne si l'Alliance Atlantique et la première et principale garantie de sécurité et du maintien de la paix en Europe si l'or sur le danger de la guerre se profile en Europe, le réflexe instinctif de protection et de se tourner vers l'OTAN, alors cela veut dire que l'Union n'a pas encore réussi à devenir ce que nous attendons d'elle les faits le démontrent de défense européenne, on est à ses balbutiements, l'armée européenne n'existe pas en dehors de quelques débats qui débouche sur quelques dans ta tentative administrative d'un régiment franco-allemand et de quelques essais infructueux sur le terrain, comme cela a été avec le la force Takuba que le président de la République nous avait vendu comme le début visible de cette armée européenne relayée ici même par le 1er ministre et la ministre des armées, la coopération européenne en matière de défense et concrètement la plupart du temps issue d'accord directement pris entre pays concernés, à ce stade, l'armée européenne ressemble à une armée de papier, mais les pluies vont Sheba avec des flèches et des pointillés décidé comme il faut voir des dons en face des fonctions ne feront jamais une armée opérationnelle sur le terrain, capable de conduire des missions et encore moins dans le cadre d'un combat défensif à haute intensité. Il ne s'agit pas de jeter ici là Pierre mais simplement de constater où nous en sommes réellement, nous avons encore beaucoup de travail avant que l'Union européenne soit en capacité de se défendre seul, en l'état, les choses sont claires : la défense européenne n'existe pas et l'armée européenne, si elle existe, ce n'est qu'au sein de l'OTAN, cette année, cette armée n'est donc pas seulement européenne mais inscrit dans un cadre plus large et étendu dans lequel les États-Unis d'Amérique ont un rôle particulier entre membres éloignés de la famille Capitaine d'équipe est leader économique, les États-Unis eux-mêmes n'ont pas toujours la même appréciation de ce que l'OTAN, souvent ils aimeraient surtout la voir comme un espace économique leur permettant de vendre leurs matériels de défense à des partenaires privilégiés, mais il faut être le plus juste possible et aussi constaté que mis à part le drame syrien et l'absence tragique de l'OTAN en 2014 alors que la France, par la voix de son président, François Hollande était engagé avec le peuple syrien, les États-Unis ont répondu présents aux côtés des Européens à chaque fois que cela s'est avéré nécessaire dans notre histoire, l'Europe a beaucoup progressé sur le fond depuis 1945 et la fin de la sauce longue guerre mondiale néanmoins elle s'est peut être trop contenté d'élargissements successifs depuis la chute du mur de Berlin sans se reposer la question de son projet de fonds et des moyens engagés dans le domaine de la défense, le retard est gigantesque entre les intentions les réalisations et les nécessités actuelles et futures, enfin cette double demande d'adhésion de la Suède, de la Finlande nous oblige à questionner le positionnement de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie, la guerre en Ukraine se poursuit avec son lot de haine et de misère, mais cette guerre, la Russie ne pourra pas la remporter l'Union européenne a et aura toujours des frontières communes avec ce pays qui est aussi un membre à part entière de la grande histoire de l'Europe, par delà le vote de ce jour, par delà les adhésions de la Finlande, de la Suède à l'OTAN nous devons aussi poser et répondre à la question de l'équilibre de de relations avec la République fédérale de la, de Russie, dès lors qu'elle aura cessé son agression et rappelé l'ensemble de ses troupes dans son espace territorial pour tout cela, le groupe socialiste soutient bien entendu la demande d'adhésion de la République de Finlande et du royaume de Suède, je vous remercie. Merci. Je donner la parole, notre collègue Joëlle Garriaud-Maylam pour le groupe des Républicains. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, c'est un honneur, mais surtout une joie pour moi en tant que vice-présidente de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et présidente du groupe des élus de droite et de centre-droit dans cette assemblée de participer à ce débat sur le projet de loi autorisant la ratification du protocole au traité de l'Atlantique nord sur l'accession de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, c'est aussi une fierté que la France soit parmi les premiers pays membres de l'alliance euro-Atlantique à être en mesure de le ratifier, dans des délais particulièrement courts, cela n'avait pas été le cas dans le passé et la France, par exemple, avait été l'avant-dernier pays à ratifier le projet de loi relatif à l'adhésion de la Macédoine du Nord à l'OTAN, dont j'étais le rapporteur ici au Sénat après un processus particulièrement long, aujourd'hui nous sommes le 19ème États entamé une procédure de ratification parlementaire et je compte sur vous, madame la ministre, pour pousser l'Assemblée nationale à suivre l'exemple du Sénat et à adopter ce projet de loi, le plus vite possible, le 18 mai dernier, la Suède et la Finlande déposer officiellement leur demande d'adhésion, 10 jours plus tard, à l'occasion de la réunion de printemps en Lituanie, de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, le président du Parlement, de Finlande Matif femme Hanane et celui du Parlement, de Suède, Andreas Norlén était venu à Vilnius nous demander de soutenir leur candidature à l'OTAN approuvé, nous avait-il dit, par plus de 80 % de leur population, nos parlementaires autant présent les avons assuré de notre total soutien et de nos efforts pour que cette adhésion soit ratifié dans les meilleurs délais cette adhésion est une impérieuse nécessité car l'histoire, vous le savez tous mes chers collègues, s'est accélérée et a pris une tournure dramatique le 24 février dernier avec l'attaque brutale et injustifiable de l'Ukraine, pays souverain, indépendant et démocratique par une Russie violent tous les principes de base de la coopération internationale et causant dévastation mort et souffrance crises humanitaires, et Ali m'enterre avec d'énormes répercussions à l'échelle de la planète puisque l'ONU estime à 255 millions les personnes pouvant souffrir de famine dans le monde, suite à cette guerre, il nous fallait être à la hauteur de l'histoire et c'est une grande satisfaction de voir que tous les pays européens, petits ou gros, se sont retrouvés pour s'engager dans l'aide à l'Ukraine, bien que celle-ci ne faisait pas partie de l'OTAN et ne pouvait donc prétendre à son aide directe sur le territoire, cette solidarité s'est affirmé lors du sommet historique de Madrid et 30 juin et 1er juillet dernier qui a vu l'unanimité de nos pays membres en faveur de cette édition, j'ai beaucoup entendu critiquer la Turquie mais je voudrais souligner ici le travail positif des parlementaires turcs, membre de l'Assemblée parlementaire a le temps pour aider à l'accord turcs lors du sommet de Madrid mais comment aurions-nous pu refuser cette demande d'adhésion de la Finlande et de la Suède, 2 pays qui partagent un car nos valeurs démocratiques des pays avec lesquels nous coopérons depuis des décennies qui ont participé à nos efforts de guerre dans les Balkans en Afghanistan Syrie mail Sahel : Mali et accueille des exercices militaires autant sur leur territoire, c'est un honneur qu'ils nous font de vouloir rejoindre notre alliance et c'est aussi une démarche d'un grand réalisme alors qu'ils étaient jusqu'à présent, attaché au plus confortable, mais un peu utopique, principe de neutralité, c'est aussi un immense service qui nous rentre dans le cadre des nouveaux enjeux stratégiques et de la défense de la paix dans toute la région, pas seulement autour de la Baltique ah c'est une dynamique vertueuse et ils nous apporteront leur expertise en termes de résilience, mais aussi leurs capacités militaires, cela a été dit Voltaire avait écrit que l'humanité n'avait jamais connu la paix seulement des entre 2 guerres, avec le temps, à Lyon, ce qui a fait ses preuves en tant que facteur de paix et de stabilité, cet entre-deux guerres a duré plus de 70 ans et notre devoir et pour les générations futures, d'éviter l'extension du conflit russo-ukrainien pour maintenir la paix en Europe avec la Finlande et la Suède, nous serons tous plus plus forts et ce sera aussi un signal fort vis-à-vis de l'agresseur russe seul accroîtra notre défense collective, ce sera aussi une protection pour ce pays, puisque l'article 5, cela a été rappelé défini, vous le savez, qu'une attaque contre l'un de nos pays est une attaque dirigée contre tous nos pays qui veut la guerre par la guerre est un principe qui a été une constante géopolitique et pour conclure, alors que la France, cela a été rappelé, a toujours été d'une grande prudence lorsqu'on parle d'élargissement j'estime aussi à titre personnel, que le Parlement a le devoir d'être un peu un aiguillon du gouvernement, surtout surtout quand il s'agit de la défense de nos peuples et c'est pourquoi je voudrais dire combien il me semble essentiel d'essayer d'être d'aider à l'adhésion d'un autre pays ami de la France, la Géorgie acquis cette adhésion a été promise depuis des décennies et qui méritent d'y entrer par ces réformes, hein, et parce que ce serait essentielle pour sa sécurité, comme je l'avais souligné dans un rapport de 2014 à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, adopté à l'unanimité, mais malheureusement non suivies au sommet du Pays de Galles de 2014 merci. Merci, ma chère collègue. Nous allons passer, si vous le voulez bien discussion des articles. Article 1er

Avis contraire. Abstentions. Les abstentions. Il est adopté. Article de. Pas de demande pas demande d'explications de vote je le soumets à votre approbation. Ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire. Abstention : il est adopté. Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par la Commission, par le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste et par le groupe, les indépendants, République et Territoires sur l'ensemble du projet de loi avant de procéder au vote, y a-t-il des demandes d'explications de vote. Je n'en vois point du protocole au traité de l'Atlantique, mort d'Atlantique nord sur l'accession du royaume de Suède. Le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos.

Résultat du scrutin numéro 124 sur l'ensemble du texte contre tenue de l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs aux groupes politiques et du notifié à la présidence, nombre de votants 348 nombre de suffrages exprimés 340 pour l'adoption 323 contre 17, le Sénat a donc adopté. Mes chers collègues, je vais maintenant lever la séance, notre prochaine séance aura lieu le mardi 26 juillet à 14 heures 30 pour l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne, la séance est levée.